La séance est reprise. Nous poursuivons l'examen du projet de loi, modifié par lettre rectificative, d'orientation des mobilités.

fait davantage écho aux enjeux de solidarité à la fois sociale et territoriale, qui sont un des fondements du projet de loi. Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable. Je mets

à M. Frédéric Marchand, sur l'article. Comme le rappelle éloquemment le laboratoire des mobilités inclusives, « pour les populations fragiles, tout est plus loin, plus cher et plus lent. [ ...] La faiblesse de leurs revenus entame leur capacité de mobilité. Et, comme un cercle vicieux, ces freins contribuent à leur tour à les maintenir dans leur précarité. » Alors qu'une partie de l'emploi tend à se concentrer dans les métropoles et qu'une bonne mobilité n'est souvent qu'un simple prérequis à l'embauche, permettez-moi d'ajouter que les populations les moins mobiles aujourd'hui sont les populations fragiles de demain. La mobilité, nous le savons, c'est l'accès à l'emploi, le droit de mener une vie personnelle épanouie et la possibilité de rendre visite à ses proches, de profiter de la vie culturelle de son territoire, de voyager. La mobilité du quotidien, c'est la liberté au fil des jours. À cet égard, la grandeur des acteurs publics est de réduire la distance qui éloigne nos concitoyens de leurs droits. Voilà ce qu'est la mobilité inclusive. L'article 6 dispose que les autorités organisatrices de la mobilité offrent un conseil en mobilité pour les personnes les plus fragiles. Il permet ainsi une meilleure information sur les solutions de mobilité, un conseil spécifique pour les publics les plus éloignés de la mobilité et une personnalisation des dispositifs par le versement d'aides individuelles. Sur l'initiative du rapporteur, nous sommes allés un peu plus loin en commission, un principe de coordination de l'action des différentes parties prenantes sur ce sujet. Cette coordination est indispensable, dans un domaine faisant déjà l'objet de nombreuses interventions, en vue d'assurer la cohérence des dispositifs existants et à venir.

ce qui était très attendu par les acteurs. Je propose de préciser ce principe en introduisant un plan d'action commun en faveur de la mobilité solidaire, ayant pour vocation d'expliciter les actions menées par les différents acteurs. Ce plan déclinerait ainsi le principe de coordination figurant dans la loi. Il serait élaboré à l'échelle d'un bassin de mobilité pour regrouper les problématiques du quotidien en matière d'accès à l'emploi, au service public, à la santé, à l'éducation et à la formation. serait placée sous la responsabilité conjointe de la région et du département, au titre de leur rôle majeur de coordination en matière, respectivement, d'organisation de la mobilité et et de solidarité. La région interviendrait aussi en tant que responsable du développement économique. Ce plan associerait les acteurs de la sphère sociale accompagnant au quotidien les personnes les plus fragiles.

vise à mieux situer la compétence « mobilité solidaire » dans la liste des compétences des autorités organisatrices de la mobilité locales et régionales.

Il s'agit d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. Le rapport souligne que, selon l'étude d'impact du projet de loi, 7 millions de Français seraient concernés par des problèmes d'accès à la mobilité. Ces difficultés de déplacement sont identifiées comme l'un des principaux obstacles à l'insertion et à l'accès à l'emploi.

aux lieux d'aide alimentaire et aux soins dispensés gratuitement dans certains hôpitaux, dans la recherche d'un hébergement ou d'un logement et dans de nombreuses démarches administratives permettant d'accéder aux droits et à l'insertion.

des seniors et des jeunes. En effet, plusieurs études récentes démontrent que ces tranches de la population connaissent des difficultés de déplacement spécifiques : les seniors seraient 5 millions à subir des freins pour sortir de chez eux au quotidien, tandis qu'un tiers des jeunes de 18 à 24 ans

prégnante s'agissant des seniors, pourtant bien souvent en situation de particulière vulnérabilité. La conséquence de cette situation est la difficulté d'accéder

pour les personnes en situation de handicap. Les ajouts prévus par le projet de loi permettront de diversifier les aides à la mobilité. L'amendement n'est donc pas nécessaire : nous en sollicitons le retrait. nous en sollicitons le retrait. L'article 6, consacré à la mobilité solidaire, vise des publics confrontés à des difficultés sociales ou économiques. En conséquence, il n'est pas opportun de faire référence de manière très générale à la mobilité des seniors et des jeunes,

Babary propose d'ajouter les apprentis dans la liste des personnes à accompagner, d'une part parce que les jeunes en apprentissage n'ont pas nécessairement l'âge d'avoir le permis de conduire, d'autre part parce que les déplacements s'organisent autour de deux destinations : le lieu d'étude et le lieu de travail. Le développement de l'apprentissage en France étant une priorité, il est nécessaire de se donner les moyens de mettre en place cet accompagnement. Quel est l'avis de la

Sincèrement, c'est un premier pas très positif, qui va dans la bonne direction, mais cela reste insuffisant pour les personnes accompagnatrices. Nous proposons donc que les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur bénéficient de la gratuité. Notre amendement va à l'encontre des modifications apportées par la commission, qui a adopté une rédaction restrictive pour les personnes concernées par les mesures tarifaires spécifiques. En conditionnant le bénéfice des tarifs spécifiques aux personnes porteuses de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion, de la mesure aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et on écarte 1 million de personnes en situation de handicap. Cette distinction entre personnes en

de dispositifs tarifaires. Pour notre part, nous refusons de sélectionner les personnes selon le niveau de leur handicap, tout comme nous refusons de sélectionner les personnes selon leur condition sociale. Le droit au transport s'applique à toutes les personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la gratuité des transports pour tous

par l'amendement n° 148 n'est pas nécessaire. Il reviendra à chaque AOM de déterminer les conditions tarifaires dont bénéficieront les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.

Il est certain que c'est cette mention qui justifie le plus le recours à un accompagnateur. Néanmoins, celle-ci est délivrée sous des conditions strictes- le taux d'incapacité doit être supérieur à 80 % -, et certaines personnes titulaires d'autres mentions peuvent avoir besoin d'un accompagnateur.

en particulier les demandeurs d'emploi ou les personnes éloignées de l'emploi. On le sait, leur insertion dans l'emploi reste conditionnée aux politiques de déplacements : c'est notamment le cas des Français vivant dans les territoires ruraux qui doivent se rendre dans les centres urbains, lesquels concentrent les emplois. Cela nous apparaît être un élément fondamental de l'inclusion sociale. Par ailleurs, il faut également répondre aux besoins de déplacements des personnes âgées, qui sont particulièrement exposées au risque de l'isolement social et de la solitude. Là aussi, nous le savons, la mobilité constitue un élément fondamental d'inclusion

car le code des transports prévoit déjà une tarification sociale en fonction d'un critère de revenu. Par ailleurs, l'article 6 du projet de loi permettra aux AOM de développer les services de conseil et d'accompagnement aux personnes en difficulté sociale,

en le complétant et en corrigeant une erreur d'insertion de la disposition dans le code des transports. La plupart des transports à la demande spécialisés dans le transport des personnes handicapées prévoient une procédure lourde, avec d'importantes contraintes : obligation de résidence, établissement

également demandée par le Défenseur des droits. En outre, la notion de « personne à mobilité réduite » est plus large que le public coeur de cible de ces services. Il est donc nécessaire de préciser que cette double simplification s'appliquera aux seules personnes handicapées et personnes à mobilité réduite titulaires d'une carte mobilité inclusion présentant un handicap de plus de 80 %.

En l'absence de mécanisme dérogatoire pour l'aménagement de places dédiées à l'implantation de bornes électriques, l'exigence prévue à l'alinéa 6 de cet article risque de freiner l'implantation de places aménagées de bornes électriques, qu'elles soient accessibles ou non. Pour éviter cet effet contre-productif, cet amendement vise à imposer un aménagement aux normes d'accessibilité des places pré-équipées ou équipées de bornes électriques au sein des seules aires de stationnement, en dehors des emprises de voirie dédiées à la circulation, dans lesquelles dans lesquelles l'aménagement de telles places ne soulève pas d'impossibilité technique récurrente. serait redondante avec l'article 23, qui prévoit une accessibilité des places dotées de bornes de recharge dans les aires de stationnement. La navette parlementaire permettra peut-être de répondre à la préoccupation exprimée, mais, à ce stade, nous préférons maintenir le dispositif initial, sauf à le vider de toute portée. En conséquence, l'avis est défavorable. Quel est Quel est l'avis du Gouvernement ? En restreignant l'accessibilité des bornes de recharge aux seules places situées dans des aires de stationnement, et non plus en voirie, l'amendement ne garantit plus le libre accès à un service public. Or le Gouvernement souhaite garantir la mobilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et leur accès au service public de recharge électrique. Il faut donc que les places en voirie disposant de bornes leur soient également accessibles. L'avis est défavorable. Je mets aux voix l'amendement n°

Jocelyne Guidez. Au vu de la mise en accessibilité progressive des réseaux de transports publics et eu égard au rôle de la région comme chef de file, l'enjeu consiste à rendre visible ce qui a été rendu accessible. En effet, la date ultime pour l'élaboration des schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée étant le 26 septembre 2024, il s'avère nécessaire, d'une part, de valoriser les actions entreprises par les autorités organisatrices de la mobilité, et, d'autre part, de permettre aux personnes âgées

chaque fin de période intermédiaire de mise en oeuvre des schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée transmis par les autorités organisatrices aux préfets. L'adoption de ces amendements conduirait à créer une nouvelle obligation administrative à la charge des régions,

madame la ministre,

des moyens de mobilité, encore faut-il que des solutions de mobilité existent ! Les voyageurs sont demandeurs, en priorité, de plus de transports, et non de gratuité. Si plusieurs collectivités territoriales

leurre le passager sur le coût réel du transport. Dans une note publiée en septembre 2018, le Commissariat général au développement durable constate que, malgré la croissance régulière des coûts d'exploitation des transports urbains, la part du coût supportée par l'usager ne cesse de s'éroder depuis quinze ans, alors que la contribution des collectivités publiques augmente. Si le coût total du transport urbain a crû de 5,2 % en moyenne annuelle de 2000 à 2015, la contribution des usagers au financement des transports en commun ne cesse, elle, de décliner. Ainsi, en 2015, les usagers supportaient 12 % du coût du transport urbain dans les réseaux de province dépourvus de métro ou de tramway, 20 % dans ceux équipés de métro ou de tramway et 38 % en Île-de-France.

Le code des transports prévoit déjà une exigence générale d'efficacité économique et sociale de la politique tarifaire. J'ajoute qu'une mission d'information sur le sujet vient d'être créée au Sénat et qu'elle pourra formuler des propositions concrètes.

seuls contribuables, favoriser une politique de report modal et de fidélisation des usagers, garantir le droit aux transports pour tous. À ce titre, je suis convaincue que la gratuité n'est pas forcément la meilleure solution ; elle l'est même rarement. La mise en La mise en place de tarifications solidaires est une solution beaucoup plus intéressante. Pour autant, il importe de respecter la liberté des autorités organisatrices de transport en matière de politique tarifaire, au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales, auquel votre assemblée est, je

Monsieur le président, madame la ministre,

amendement prévoyait que les autorités organisatrices des mobilités en outre-mer puissent mettre en place toute forme d'aide ou de dispositif afin d'assurer la continuité territoriale sur l'ensemble de

en matière économique et environnementale, mais aussi en termes d'équité territoriale et sociale, il est urgent, pour nos territoires insulaires d'outre-mer, et singulièrement la Guadeloupe, qui est un archipel, d'organiser un service public des mobilités,

Si le présent projet de loi n'aborde pas les questions de transport aérien, il met en avant le mot « mobilité » ; c'est sur ce mot, précisément, que porte le message de Robert Laufoaulu. Comment peut-on parler de mobilité lorsque deux îles distantes l'une de l'autre, mais aussi, et surtout, éloignées des États voisins et des autres territoires français du Pacifique sont soumises au bon vouloir d'une compagnie aérienne en situation de monopole, avec tout ce que cela implique en termes de fixation de prix, d'horaires et de nombre de liaisons ?

Le président François Hollande, en visite sur le territoire, avait pris conscience du problème et s'était engagé en faveur d'une desserte Fidji. Le lancement d'un appel d'offres a été décidé ; toutes les entraves ont été mises en oeuvre pour que ce projet n'aboutisse pas. À qui profitent ces tristes manoeuvres ? Le bureau d'études chargé de rédiger l'appel d'offres pour la desserte de Wallis s'est arrêté à Nouméa. Il ne s'est même pas rendu à Wallis-et-Futuna. Pourquoi ? Les Fidjiens avaient signifié leur intérêt pour une desserte de Wallis-et-Futuna. On leur a fait comprendre que cela posait problème. Qui est ce « on » ? Parlons aussi de la desserte entre les deux îles de Wallis et de Futuna. La notion de vétusté n'existe pas en matière civile. Le territoire a dépensé de l'argent, chaque année, pour l'entretien et le remplacement des pièces de l'avion. Quelles sont les raisons de son retrait et de sa vente programmée ? Madame la ministre, la continuité territoriale et la mobilité sont des notions qui doivent également concerner Wallis-et-Futuna. Une mission est envisagée pour le mois d'avril, afin de faire le point sur la situation et avancer des propositions de sortie de la convention actuelle. Les Wallisiens craignent que cela n'aboutisse qu'un nouveau rapport, et rien de plus ! Comment être assuré que ces travaux pourront déboucher sur des résultats, tant espérés, mais jamais atteints ? Il ne pourra jamais y avoir de développement de Wallis sans désenclavement aérien, et les Wallisiens ne peuvent être ainsi à la merci des intérêts des autres. Ils ne veulent pas continuer à subir leur destin ; ils veulent être acteurs de leur développement. Wallis-et-Futuna et ses habitants comptent sur le Gouvernement pour s'engager en ce sens. La parole

Un appel d'offres avait été lancé en juin 2017, avec deux lots, portant l'un sur les services intérieurs, l'autre sur une liaison aérienne internationale entre Wallis et Nadi. Wallis et Nadi. Il a dû être déclaré infructueux, s'agissant du second lot, le niveau de subvention demandé par les candidats excédant très largement le budget prévisionnel. Quant à la desserte intérieure, l'augmentation du nombre de fréquences régulières hebdomadaires n'a été rendue possible qu'au prix d'un soutien financier plus important de l'État et du territoire. Dans ce contexte, l'ensemble des parties à la délégation de service public pour les services intérieurs- l'opérateur, l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna et ses services, ainsi que la direction générale des outre-mer -sont convenus de redéfinir les termes organisationnels, opérationnels et financiers, au plus tard le 30 juin 2019. Un groupe de travail a été mis en place à cette fin. Il a débuté ses travaux au début de l'été 2018.

Nous avons donc, avec madame Girardin, demandé à ce qu'une mission d'inspection vienne en appui et contribue aux réflexions de ce groupe de travail. J'ai bon espoir que la complémentarité ainsi créée permette de trouver des voies d'amélioration pour l'ensemble de la desserte du territoire, qu'elle soit aérienne ou maritime,

Cela favorisera la réalisation de plans de mobilité dans les outre-mer, aux fins d'identifier avec précision les besoins et les évolutions de la mobilité dans ces territoires. Quel est l'avis de la

des territoires ultramarins, et donc de déterminer si la proposition est adaptée à ces spécificités ou s'il est préférable de maintenir le régime existant. Dès lors, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement. Quel est

moins dépendants des importations d'hydrocarbures et à tirer profit des ressources naturelles et technologiques disponibles, afin de développer l'utilisation de véhicules propres.

relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier des personnes. L'exemption des DROM de l'application du dispositif de la LOTI visait à prendre en compte les difficultés en matière de transport collectif en outre-mer, liées aux distances séparant villes et villages. cette exemption ne se justifie plus, notamment en Guadeloupe : depuis 2016, le syndicat mixte des transports a déployé un réseau couvrant efficacement le périmètre des communes incluses dans le plan de déplacement urbain. Elle a désormais pour seule conséquence une concurrence déloyale pour les taxis d'outre-mer.

transport public particulier des personnes, le législateur avait souhaité exclure les départements ultramarins de l'application de certaines dispositions, compte tenu des spécificités locales en matière d'organisation des services de transport. Dans le temps imparti, nous n'avons pas pu réexaminer la question pour déterminer s'il est nécessaire de revenir sur ce choix.

de fournir des services occasionnels de transport particulier de personnes dans les agglomérations des DROM à forts flux touristiques et économiques. Je voudrais rappeler que la disposition de la loi Grandguillaume

Ensuite, il me semble que le tissu économique des territoires ultramarins est fragile et que cette disposition pourrait mettre en difficulté un très grand nombre d'entreprises, qui seraient dans l'incapacité de basculer dans le régime VTC, plus contraignant. L'expérience du basculement en métropole montre toute la complexité d'un tel changement. Enfin, une telle mesure ne peut être adoptée sans une évaluation des enjeux, sans une concertation préalable avec les acteurs et, en tout état de cause, sans prévoir une période de transition minimale. Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.

Cet amendement vise à mieux définir la politique de continuité territoriale outre-mer,

commission ? Dans la mesure où la politique de continuité territoriale vise l'outre-mer dans son ensemble, y compris les territoires composés de plusieurs îles, cette précision serait d'une portée limitée. À l'inverse, si elle vise à confier à l'État une mission relevant des collectivités,

rédigé, vise à étendre la politique nationale de continuité territoriale à des services de transport intérieur aux collectivités. Son adoption reviendrait à prévoir une intervention de l'État

C'est pourquoi la commission a adopté cette motion, tendant à proposer au Sénat de déclarer ces amendements irrecevables. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est très claire quant à l'inconstitutionnalité de tels amendements. De surcroît,

Nous ne sommes pas opposés par principe à cette démarche, qui participe de la transparence de l'organisation des services publics et favorise la mise en oeuvre des nouveaux services. Nous sommes en revanche plus circonspects sur les conditions de réutilisation de ces données publiques.

Aujourd'hui, nous voyons bien, d'ailleurs, la difficulté qu'ont les pouvoirs publics à faire respecter par les Gafam les règles nationales, notamment en matière d'impôts. Nous ne souhaitons donc pas alimenter par ce biais la machine à évasion fiscale. Sur le fond, nous craignons non seulement qu'étendre l'obligation d'ouverture des données aux données dynamiques ne crée une charge très importante pour les autorités organisatrices et leur opérateur, mais également que cet investissement soit, comme nous le disions, capté par les GAFAM, qui pourront en disposer gratuitement pour développer des applications payantes et lucratives. Pour cette raison, nous souhaitons la suppression de la mise à disposition des données dynamiques. En effet, tel qu'il est rédigé, le présent article va au-delà des obligations et du règlement européen de 2017. Celui-ci impose uniquement que le point d'accès contienne au moins les données statiques sur les déplacements et la circulation, ainsi que les données historiques concernant la circulation des différents modes de transport, y compris les mises à jour des données. Les États conservent donc pleinement une marge de manoeuvre pour imposer ou non l'accès aux données dynamiques. Nous proposons de limiter l'ouverture des données aux seules données théoriques, laissant le soin aux autorités organisatrices d'aller plus loin dans l'offre

Quel est l'avis du Gouvernement ? Le règlement européen de 2017 sur l'information multimodale contient une partie consacrée aux données en temps réel et laisse à la discrétion des États la décision d'ouverture de ces données. Demander l'ouverture des données en temps réel n'impose pas que ces données doivent être créées, mais seulement qu'elles doivent être rendues accessibles si elles existent. Or il y a une forte attente des voyageurs pour une information en temps réel portant notamment sur les véritables horaires des transports publics et sur les incidents -par exemple les bouchons sur les routes. Par ailleurs, en l'absence d'ouverture des données des autorités organisatrices, les grands acteurs du numérique, grâce à leur notoriété, à l'importance de leurs moyens ou de leur audience, seront seuls en mesure d'obtenir ces données ou de les créer eux-mêmes sur l'ensemble du champ de la mobilité. L'ouverture des données permet donc d'améliorer le jeu de la concurrence et de l'innovation. Toutes les entreprises ont accès aux données et la concurrence joue pour des services de meilleure qualité pour les usagers. Je suis défavorable à cet amendement.

Loin de moi l'idée de renforcer les préjugés sur les moyens de transport toujours en retard, mais, en ce qui concerne l'ouverture des données, force est de constater que beaucoup reste à faire. Si les conditions d'indemnisation en cas de retard sont publiques, n'est pas publique la base de données des retards, à partir de laquelle l'opérateur va appliquer son barème d'indemnisation.

Le voyageur, notamment étranger, sera alors remboursé, ce qui ne pourra que faire progresser le recours aux modes de transport collectif et la confiance à leur égard. Ces données existent déjà. Les ouvrir renforcerait les droits des voyageurs

Cela aboutirait à une très importante simplification de formalités pénibles pour le voyageur. La levée de ce type de barrières facilitera le recours aux modes de transport collectif massifié, dont les vertus environnementales sont bien connues, non seulement pour la mobilité du quotidien, mais aussi pour les voyageurs internationaux, souvent non francophones.

de ces amendements d'aider les voyageurs à faire valoir leurs droits en cas de retard, mais la rédaction proposée ne limite pas l'ouverture des données à ce cas et pourrait concerner un champ très large de données pouvant par ailleurs avoir une forte valeur économique pour certains acteurs. En outre, ces données de retards constatés ne figurent pas dans la liste des données à ouvrir définie par le règlement européen. Pour des questions de clarté de la loi, ce sujet devrait donc être traité dans une partie séparée de l'article L. 1115-1

Madame la ministre, et, sur décision des États, les données dynamiques. Les personnes tenues d'ouvrir leurs données à ce titre sont donc les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructures et les autorités organisatrices. Cet amendement vise à étendre cette obligation aux dispositifs mobiles et connectés. Je partage tout à fait l'ambition que ces données

L'article 9 confie aux métropoles et aux régions le soin d'animer les démarches de fourniture des données au point d'accès national. Ces AOM doivent s'assurer de la conformité des données fournies aux normes fixées par le règlement européen. L'article prévoit que les régions assument cette tâche sur la partie du territoire régional qui ne relève pas d'une métropole et autorise les métropoles à utiliser ces données sur leur seul territoire administratif, alors que leur rayonnement en termes de mobilité dépasse très largement

fournir ce service de données au-delà de leur seul périmètre administratif, dès lors que la région est d'accord, nous semble représenter un véritable progrès.

complétant la directive du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux. Ce règlement fixe les modalités de centralisation des données de mobilité, afin de mieux appréhender les usages et besoins sur chaque territoire et d'améliorer l'information de l'usager, pour lui offrir plusieurs solutions de mobilité et favoriser ainsi la multimodalité. Il prévoit également une mise à disposition de ces données pour utilisation et traitement par des opérateurs tiers, le cas échéant par le biais d'un accord de licence. S'il convient de favoriser l'innovation en permettant l'étude de ces données, il est également essentiel, d'une part, de garantir la confidentialité des informations transmises par chaque opérateur aux autorités, afin que la stratégie de déploiement d'un opérateur donné ne puisse être analysée par ses concurrents directs, et, d'autre part, de s'assurer que l'accès aux données agrégées ne permet pas à un opérateur de construire une situation dominante sur le marché.

demain une position concurrentielle dominante. ? Plusieurs éléments paraissent discutables s'agissant de ces amendements très proches. En premier lieu, l'ouverture des données, telle qu'elle est prévue par le règlement, ne porte ni sur des données à caractère personnel ni sur des données stratégiques et donc confidentielles.

Jean-François Longeot. La quatrième révolution industrielle repose sur une économie de la donnée. Nous devons sortir de notre inertie en la matière et nous engager résolument dans cette révolution. Il y va de notre souveraineté. Mais notre rôle est également de nous assurer que ce nouveau pétrole de l'économie mondiale soit au service de l'intérêt général, qu'il soit un gage des politiques publiques de mobilité construites par des autorités organisatrices de la mobilité.

En effet, les conditions d'utilisation des données actuellement disponibles sur le point d'accès national sont exclusivement définies par la licence ODBL, celle-ci ne permettant ni de suivre les usages des jeux de données ni de s'assurer de leur compatibilité avec les politiques publiques de mobilité. Les autorités organisatrices des mobilités doivent pouvoir proposer leur propre licence ou recourir aux licences existantes, dès lors qu'elles ne limitent pas les possibilités de réutilisation et ne sont un frein ni à l'innovation ni à la concurrence. La seconde partie de l'amendement vise en effet à identifier les utilisateurs qui contreviendraient aux conditions de réutilisation des données fixées dans le cadre de la licence. Le point d'accès national pourra procéder à une mise en demeure ou à une suppression de l'exécution des modalités de mise à disposition des données à l'encontre de l'utilisateur dont l'usage des données serait contraire aux politiques publiques de mobilité construites par l'AOM. Quel La préoccupation des auteurs de cet amendement me paraît pleinement légitime : il s'agit notamment d'autoriser les AOM à définir des conditions de licence leur permettant de s'assurer du respect de leurs politiques de mobilité par les réutilisateurs de données. Cela paraît cohérent, toutefois ils proposent de confier au point d'accès national un rôle que le projet de loi confie à l'Arafer.

du Gouvernement ? Je partage tout à fait le souci de définir des règles d'accès aux données équitables et ne restreignant pas la concurrence. Le dispositif mis en place avec le point d'accès national consiste, pour ce qui concerne le contenu des licences de réutilisation, d'une part à s'appuyer sur la règle générale du règlement européen- les conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation -, d'autre part à unifier les licences afin de fluidifier l'accès aux données. L'un des principaux bénéfices du point d'accès numérique pour l'écosystème de la mobilité est l'harmonisation des conditions d'utilisation des données sous licence ODBL, gage d'ouverture réelle, neutre, sans discrimination ni biais.

En outre, la procédure de suppression de la fourniture des données à un réutilisateur qui ne respecterait pas ces règles figure déjà à l'article 9, alinéa 31, du projet La procédure est confiée à l'Arafer, parce qu'il semble préférable que ce soit une autorité indépendante qui puisse décider de façon sûre d'une telle mesure conservatoire, ce qui protège le producteur des données

l'amendement n° 151. Les garde-fous prévus par le texte, malgré les efforts du rapporteur, pour faire payer les utilisateurs de données seulement au-delà d'un certain seuil de requêtes

Or les sociétés qui exploitent les données fournies ont jusqu'à présent mis en place des contre-feux pour rester en deçà de ce seuil, notamment grâce à un changement d'adresse IP.

des dizaines de millions d'euros. Il faut aussi des serveurs suffisamment puissants pour supporter un grand nombre de requêtes. Un coût d'exploitation, ensuite : il faut notamment payer les personnels de régulation qui, en adaptant l'offre en temps réel, génèrent ces données et il faut payer la maintenance des applications. L'Union des

-veulent utiliser ces données pour faire du profit, il est logique de les faire payer dès la première requête en intégrant ces deux éléments. Il s'agit, je le rappelle, d'une mesure compatible avec le règlement européen de 2017. Nous proposons donc que l'utilisateur s'acquitte d'une compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.

est d'éviter les situations de rente et de permettre l'innovation. Elle me paraît satisfaisante. L'avis est donc défavorable, même si l'on peut considérer effectivement qu'il sera délicat de définir des critères insusceptibles d'être contournés.

Néanmoins, remettre en cause la gratuité pour les petits utilisateurs ne me semble pas opportun : cela pourrait freiner l'innovation que l'on peut attendre de la part de start-ups ou d'acteurs à faibles moyens.

pour éviter tout risque de contournement du seuil de gratuité. Pour les acteurs qui ne respectent pas les règles, je rappelle la procédure de suppression de fourniture de données, que j'ai mentionnée à l'occasion de l'examen de l'amendement précédent. Je demande le retrait de ces amendements ; sinon, l'avis sera défavorable.

pour tous les usagers éligibles aux tarifications sociales. Il s'agit de garantir une information transparente, accessible et de qualité, notamment au sujet des politiques tarifaires en vigueur. Les régions et les métropoles devront à disposition des usagers un portail numérique d'information, ainsi que des dispositifs non numériques, dédiés aux aides financières individuelles liées à la mobilité, en concertation avec l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes sociaux et les opérateurs de transport.

En outre, il tend à imposer aux services d'information sur les déplacements de fournir des renseignements sur l'accessibilité des modes de transport. La mise à disposition d'une information centralisée sur les aides financières contribue à améliorer le recours aux aides par les personnes qui en ont besoin pour assurer leurs déplacements du quotidien. De même, il est nécessaire de fournir une information fiable relative à l'accessibilité des services. Toutefois,

ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Pour ces raisons, et afin d'éviter les redondances, je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, j'émettrai

Ce projet de loi a pour objet de faire évoluer le rôle de la puissance publique pour l'adapter au mieux à la transformation générale des transports et aux particularités locales en matière de mobilité.

Dans les territoires les moins denses, l'ouverture des données des véhicules taxis peut permettre d'améliorer l'offre de mobilité, dans la mesure où les chauffeurs travaillent principalement sur rendez-vous et ont donc un usage limité des applications en temps réel.

Une transmission obligatoire des données n'aurait pas d'impact sur l'offre déjà disponible les applications. Au contraire, si les chauffeurs étaient tenus de répondre aux demandes du registre national,

Gouvernement ? L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose déjà que le professionnel communique aux consommateurs certaines informations avant la conclusion d'un contrat de vente.

arrêtés de circulation qui, aujourd'hui, sont à la fois difficilement accessibles et déterminants pour le choix d'un itinéraire destiné aux véhicules lourds et de livraison. Cette information supplémentaire permettra d'optimiser la circulation de ces véhicules. En résulteront un gain de temps et un meilleur respect des prescriptions des autorités de police.

des professionnels du transport de marchandises, mais aussi d'une nouvelle contrainte susceptible de peser sur les collectivités territoriales concernées, même si elles disposent de l'ensemble des informations en question.

Le code des relations entre le public et l'administration prévoit d'ores et déjà que toute information disponible sous un format numérique doit être publiée dans un standard ouvert et aisément réutilisable.

information et billettique multimodale, afin d'offrir à l'usager un service simple et complet répondant à ses besoins pour acheter des trajets de bout en bout. Le nouvel article L. 1115-8 du code des transports serait ainsi destiné à lever les obstacles à la mise en place de services de billettique multimodale

doivent pouvoir veiller à ce que les services de billettique multimodale soient compatibles avec l'intérêt général. En ce sens, on voit bien qu'elles ont un rôle particulier à jouer. Néanmoins, afin d'assurer la robustesse juridique du dispositif garantir son caractère équilibré entre acteurs économiques, il est nécessaire de ne pas traiter de manière discriminatoire les acteurs publics et privés et d'apporter un ensemble de garde-fous aux services de mobilité. Il ne faudrait pas que la mise en oeuvre des dispositions de cet article aboutisse à les désintermédier. là, pour le Gouvernement, de deux points de vigilance particuliers. Pour ces raisons, et afin de tenir compte des orientations prises par le Sénat, j'ai relancé la démarche de concertation avec les acteurs, en vue d'aboutir à un dispositif qui permette à la fois de faciliter l'émergence de services « sans couture » pour la mobilité du quotidien de nos concitoyens,

Les usagers des services de la SNCF constatent avec regret que les personnes à mobilité réduite rencontrent des difficultés lorsque leurs voyages conjuguent l'emprunt de trains nationaux et régionaux. Par ailleurs, la multiplicité des contacts régionaux ne facilite pas la compréhension de l'organisation des transports et des voyages. Enfin, l'ouverture à la concurrence des transports ferrés,

et les interfaces entre entreprises ferroviaires pour tout ce qui a trait à la prise en charge des voyageurs. Les premiers opérateurs alternatifs pourraient arriver en 2021 : il nous faut construire un dispositif efficace

Pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter au maximum l'utilisation des différentes solutions de transport du quotidien, et donc d'améliorer l'accès à l'information sur ces solutions, ainsi

organisatrice de la mobilité, et ne couvre donc pas les liaisons entre les différents territoires de compétence des AOM. Cet amendement tend également à permettre la vente de titres de transport en dehors du territoire concerné. Ce serait, à notre sens, un facteur d'attractivité.

Par ailleurs, en vue de l'ouverture à la concurrence, il est impératif que les mêmes règles s'imposent à toutes les entreprises ferroviaires actives sur le réseau ferré national, afin de ne pas faire peser des contraintes sur le seul acteur historique. historique. Il est, enfin, important d'assurer un principe de non-discrimination entre les différents canaux de vente, de manière que les voyageurs puissent avoir un accès facilité à l'intégralité de l'offre, en toute transparence.

à l'Arafer la compétence de régulation du secteur de la distribution. Cette instance est en effet la plus à même d'apporter une réponse efficace. Toutefois, madame la ministre, seul le Gouvernement peut avancer sur ce point. L'adoption d'un tel amendement nous semble particulièrement souhaitable pour faciliter le quotidien des voyageurs et renforcer l'attractivité des modes de déplacement propres.

devront respecter un principe de non-discrimination entre les différents canaux de vente, qu'il s'agisse de filiales des entreprises de transport ou de services numériques de vente non liés à ces entreprises. Chaque canal sera en mesure de proposer à la vente l'intégralité des titres commercialisés par l'entreprise. Cette concurrence supplémentaire

L'article 11, tel qu'il est rédigé, n'ouvre pas explicitement la faculté, pour un service numérique multimodal titulaire d'un agrément, de sous-licencier cet agrément, notamment à un prestataire étranger. cette possibilité est le plus souvent exclue des contrats liant les opérateurs de transport aux services numériques multimodaux agréés. La rendre de droit facilitera l'accès au marché ferroviaire français pour certains voyageurs étrangers, sans pour autant faire courir le risque d'une dérégulation du marché ou d'une quelconque perte de contrôle de l'opérateur ferroviaire, puisque serait maintenu le principe d'une totale responsabilité de la personne agréée à l'égard de l'opérateur en cas de sous-licence.

imposer une telle solution pour l'ensemble des modes de transport sur tout le territoire, sans distinction, semble disproportionné. Je m'interroge sur les effets de la mise en oeuvre d'un tel dispositif sur la tarification des transports publics. Cela m'avait conduit à ne pas proposer un tel dispositif en commission et à privilégier une solution au bénéfice des autorités organisatrices, sous leur contrôle et sous celui des collectivités. La prudence commande donc d'émettre un avis défavorable sur ces trois premiers amendements identiques. n 38 rectifié , 811 et 841 rectifié , l'idée est intéressante, mais je remarque que le droit en vigueur les satisfait partiellement. À ce jour, en matière ferroviaire, l'autorité de la concurrence permet aux acteurs numériques d'avoir accès à la distribution à la distribution de la SNCF, en raison de la situation particulière de cette entreprise sur le marché. L'ordonnance du 12 décembre dernier permet également d'ouvrir la billettique des services ferroviaires conventionnés, en partant du principe que ces services sont dans une situation de marché particulière. Je ne suis pas certain, à ce stade, qu'il faille aller plus loin, en obligeant les opérateurs agissant sur un marché concurrentiel à respecter des obligations particulières s'ils souhaitent sous-traiter leur distribution partout sur le territoire.

Dans l'esprit du texte initial, tous les services numériques multimodaux seraient bénéficiaires de cette ouverture de l'accès à la billettique, et pas seulement les autorités organisatrices.

élargissent également l'accès aux services de billettique à tous les transports, y compris à des services librement organisés opérés à l'échelle de la France. Cela concerne les cars longue distance, mais aussi les TGV.

La concertation entre les acteurs est en cours sur les mesures qu'il conviendrait de prendre pour favoriser une billettique multimodale. Je sollicite le retrait de ces amendements.

par conséquent de la négociation entre l'entreprise de transport et le fournisseur du service numérique multimodal. Sauf à ce que ce sujet émerge comme consensuel dans les concertations, il ne semble pas nécessaire de légiférer. Je demande également le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.

au nom de mon collègue Léonhardt, vise à garantir aux habitants d'Île-de-France un égal accès à l'information dans leur utilisation des transports publics au quotidien.

Les départements de la grande couronne sont en effet presque systématiquement les derniers à bénéficier des installations les plus modernes en matière de mobilier urbain pour les transports publics, par exemple les abribus avec panneau d'information en temps réel, que l'on peut aujourd'hui observer partout dans la ville de Paris.

Le présent amendement vise donc à corriger en partie cette disparité en imposant à Île-de-France Mobilités d'élaborer un cahier des charges unique et homogénéisé, auquel seront soumis l'ensemble des prestataires avec lesquels cet établissement contracte dans ce domaine.

Madame la ministre, sur l'ensemble de ses infrastructures, s'agissant, en particulier, de l'information en temps réel dans les abribus. Je partage la volonté d'assurer une bonne information de l'ensemble des usagers, cependant il appartient à Île-de-France Mobilités, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France, de définir sa politique en matière d'information des voyageurs, y compris en termes de supports. Par ailleurs, imposer des contraintes identiques sur un territoire très vaste, sans prendre en compte des spécificités locales, paraît contraignant.

Je ne surprendrai personne en disant que nous souhaitons supprimer cet article parce que nous nous opposons au recours systématique aux ordonnances, qui prive le Parlement de son pouvoir

Mme la ministre. fait qu'il s'agit en l'espèce de préparer le cadre de déploiement du véhicule autonome. C'est évidemment un enjeu industriel majeur, et il serait tout à fait regrettable que la France prenne du retard dans ce domaine.

Nous avons été très nombreux à cosigner cet amendement proposé par M. Karoutchi, qui vise à faciliter le recours aux expérimentations de véhicules autonomes en conciliant la nécessaire souplesse, pour permettre leur essor rapide, et le respect des règles de sécurité et d'assurance, qui doivent continuer à s'appliquer. Compte tenu du lancement de la stratégie nationale pour le véhicule autonome et de la large réponse des territoires en soutien à ce développement, il convient de permettre, dans des conditions simplifiées, les expérimentations sur des itinéraires qui auront été préalablement aménagés et en constitueront le terrain de jeu. Par cohérence Par cohérence avec la mise en place des voies auxiliaires, dont l'usage doit permettre de lutter contre la congestion par des moyens qui dépendent des contextes spécifiques, l'amendement tend à supprimer une contrainte légale qui empêche, en particulier, d'encourager le covoiturage.

Il y a une autre dimension qui nous tient à coeur : l'impact environnemental du véhicule autonome, que l'on ne peut pas passer sous silence. On le sait, le développement des véhicules autonomes aura un effet majeur

Nos interrogations sont d'autant plus grandes que le Gouvernement a décidé de légiférer par ordonnance sur le sujet, par le biais de l'article 12 du projet de loi. Nous souhaitons également attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre en compte le futur le futur impact écologique de la généralisation massive des véhicules autonomes. En effet, comme vous le savez, mes chers collègues, les fameux, ces immenses infrastructures informatiques qui stockent les données numériques, ont une consommation énergétique particulièrement importante, pour ne pas dire gigantesque. En 2017, ils engloutissaient déjà près de 18 % de la consommation énergétique mondiale. On peut légitimement penser que la généralisation future du véhicule autonome aura un impact significatif sur la consommation électrique à l'échelle internationale. Il existe donc une nécessité d'information sur une technologie qui risque de se développer assez rapidement. Certes, il s'agit d'une demande de rapport

du Gouvernement ? Je partage votre préoccupation. Les véhicules automatisés destinés au transport de personnes et de marchandises pourront permettre des conduites plus fluides et des optimisations de circulation ou de parcours plus respectueuses de l'environnement. Ces technologies se développent en même temps que les nouvelles motorisations alternatives, le partage de l'usage des véhicules et la fourniture de services de transport à la demande. Les impacts dépendront largement de la façon dont les autorités organisatrices se saisiront des outils de la loi d'orientation des mobilités,

Je propose donc une nouvelle version apportant des précisions sur les finalités de l'ouverture et de la transmission des données générées par les véhicules, à la suite des échanges que j'ai eus avec M. le rapporteur et Mme le rapporteur pour avis de la commission des lois. Elle apporte les garanties attendues à l'égard des conducteurs des véhicules. ailleurs, elle intègre plusieurs propositions du Sénat, comme l'accès aux données par les autorités organisatrices de la mobilité. L'accès aux données des véhicules connectés contribuera à l'amélioration de la sécurité routière, de la gestion des infrastructures et des politiques de mobilité. C'est tout l'enjeu de ce cadre à construire. Plus précisément, l'habilitation permettra de traiter des enjeux liés à la connaissance du patrimoine routier et du trafic. Elle éclairera également les enquêtes de police judiciaire sur les accidents et les enquêtes post-accident, corrigera corrigera certains défauts de sécurité de série sur les véhicules et améliorera les algorithmes de conduite automatisée. Elle permettra aussi la réparation des véhicules avec des conditions d'accès non discriminatoires entre acteurs économiques d'un même marché, dans le respect des exigences de protection des données individuelles et de sécurité et d'intégrité des véhicules. Enfin, après agrégation, elle fournira les données de déplacement pour permettre aux autorités organisatrices de mobilité de mieux accomplir leur mission. L'habilitation que le Gouvernement sollicite me semble donc répondre aux enjeux d'avenir et comporter les garde-fous qui sont nécessaires.

des véhicules connectés et des assistants de conduite, notamment aux forces de l'ordre et aux services d'incendie et de secours. Cet article a été supprimé en commission, au motif que le champ de l'habilitation était trop large et la rédaction proposée, trop imprécise. En effet, au-delà des enjeux majeurs de sécurité couverts par cet article, le potentiel économique offert par le véhicule connecté est immense, qu'il s'agisse de la vente de ces véhicules ou du développement des services associés. Or l'accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite est aujourd'hui indispensable pour permettre de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule. Afin que cette technologie puisse bénéficier à l'ensemble des opérateurs de services, le présent amendement vise à définir les modalités et les conditions d'un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés et d'inscrire ce cadre directement dans le projet de loi. À ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d'accès semblent s'être cristallisées sont la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles, l'assurance et l'expertise automobiles, les services destinés à faciliter la gestion de flottes, la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l'alimentation en carburants alternatifs, ainsi que la création de services innovants à partir de données issues des véhicules. Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est nécessaire de fixer des conditions d'accès aux données non discriminatoires pour l'ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée. La parole

Certaines définitions sont juridiquement plus acceptables, notamment sur le véhicule connecté, et vous avez apporté des garanties sur l'utilisation des données. Comme nous le souhaitions, le nombre de destinataires de certaines données a été élargi, mon collègue en a parlé,

pour attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un scandale dénoncé à l'Assemblée nationale par le député Jean-Louis Thiériot. C'est peu connu, mais, aujourd'hui, les services de secours en intervention- pompiers, police, SAMU, gendarmerie -doivent payer leur péage comme n'importe quel usager. Pour diminuer les coûts, ces services publics ont donc pour instruction d'éviter d'emprunter les autoroutes, sauf urgence vitale avérée, ce qui, l'on s'en doute, peut avoir des conséquences dramatiques si l'on a sous-estimé la gravité de l'intervention. Or la loi de finances pour 2018 prévoit que les véhicules de secours doivent être exonérés de péage. Mais le décret d'application de cet article n'est toujours pas sorti, et les sociétés d'autoroutes n'ont pas trouvé bon de le mettre en oeuvre de leur propre chef, alors même que l'enjeu n'est que de quelques millions d'euros sur des profits annuels qui se chiffrent en milliards Interrogée sur les raisons de ce retard, l'administration a clairement répondu qu'elle refusait de publier le décret, au triple motif ahurissant que « le caractère opérationnel du déplacement est difficile à évaluer », qu'il y aurait « rupture de l'égalité » et que « les sociétés concessionnaires auraient le droit d'en obtenir le remboursement.

en ajoutant que l'accès aux données se fait « dans le respect des principes de non-discrimination et des droits garantis par le secret industriel, commercial et de propriété intellectuelle

Mme Éliane Assassi. L'article 14 tend à habiliter le Gouvernement à légiférer encore une fois par ordonnance, afin d'expérimenter des solutions de mobilité dans les zones peu denses. Ces expérimentations portent sur le covoiturage, le transport particulier de personnes et le transport d'utilité sociale.

c'est un mode de transport polluant. Cependant, nous nous opposons à la méthode employée par le Gouvernement. Il nous semble en effet que cette question mérite, comme d'autres, un débat plus approfondi, notamment dans la situation je me permets de vous rappeler que l'une des revendications des mouvements sociaux actuels est le maintien des services de proximité. Il s'agit des bureaux de poste, des écoles, des maternités, mais aussi des petites lignes de train, dont les fermetures se succèdent depuis plusieurs mois. Cet article vise à développer les moyens alternatifs à la voiture, tel que le covoiturage. Mais il existe déjà un moyen alternatif, à savoir le réseau ferroviaire. Face aux 56 lignes de train et

supérieure à ce qui se pratique aujourd'hui dans le cadre du covoiturage, ce que l'on appelle le partage de frais. Il est utile que de telles expérimentations puissent avoir lieu pour offrir des solutions de mobilité à nos concitoyens qui vivent dans les « zones blanches de la mobilité », à savoir, essentiellement, les territoires peu denses. La commission a donc émis un avis défavorable

défendu, monsieur le président. Quel est l'avis de la commission ? L'ajout proposé est très large et peu précis. Je préfère en rester à la rédaction issue des travaux de la commission, qui indique précisément les sujets sur lesquels des expérimentations nécessitant des dérogations à la loi pourront être menées dans les zones peu denses.

présenter l'amendement n° 791 rectifié. Le titre II du présent projet de loi vise à encourager les innovations en matière de mobilité. Les nouvelles solutions et nouveaux usages doivent être intégrés non seulement dans les politiques publiques de mobilité, mais également dans les outils contractuels au service de ces politiques, tels que les concessions de service public de transport. C'est pourquoi cet amendement vise à remettre aux AOM la faculté de prendre en compte ces innovations dans le secteur du transport et de favoriser de nouvelles solutions, tout en garantissant le respect des règles de la commande publique. L'amendement n° 845 rectifié n'est pas soutenu. Quel